Ces amendements ont vocation à donner aux maires des pouvoirs de modulation de la durée maximale de location des meublés de tourisme.

de délibérer pour que, dans leur ville, on ne puisse pas louer sur ce type de plateformes plus de 30 jours, 60 jours ou 90 jours,

le temps à la loi ÉLAN produire ses effets. Elle a permis d'atteindre un équilibre entre le droit de propriété et la lutte contre les pénuries de logements, en durcissant les règles applicables.

dans les zones touristiques. J'habite moi-même une commune littorale où les effets de l'activité de ces plateformes de location se manifestent.

J'entends l'argument de Julien Bargeton sur la différence entre professionnels et particuliers. Cela étant, la possibilité, pour les particuliers,

ainsi libellé : La parole est à M. Olivier Jacquin. Cet amendement vise à lutter contre les dépôts sauvages. Dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police, le maire se trouve démuni pour sanctionner le non-respect de la réglementation en la matière. La voie pénale n'est pas toujours adaptée, notamment en raison des classements sans suite, très fréquents. Elle n'apporte de surcroît aucune solution pour la réparation des dommages. La voie administrative est rarement employée alors qu'elle permet, à travers la procédure de l'exécution d'office des travaux, de remédier aux désordres La procédure administrative courante, définie à l'article L. 541-3 du code de l'environnement, s'applique à tous les manquements relatifs à la réglementation sur la gestion des déchets, depuis la décharge illégale de plusieurs hectares jusqu'au mètre cube de gravats abandonnés au bord d'un chemin. Dans les faits, elle est surtout adaptée aux procédures mises en oeuvre par les services de l'État. Introduire une procédure plus adaptée aux besoins des maires dans le code général des collectivités territoriales permettrait de distinguer la procédure pour les atteintes majeures à l'environnement, qui relèvent plutôt des services de l'État, et la lutte contre les dépôts sauvages, qui relève de la compétence des maires. Dans le cas de la lutte contre les dépôts sauvages, il est nécessaire d'intervenir assez rapidement, car l'absence de sanctions pendant une durée longue- durée longue- le temps de la procédure -confirme les contrevenants dans le sentiment de leur impunité et incite d'autres contrevenants à déposer des déchets sur le dépôt existant. C'est pourquoi l'amendement proposé inverse l'exécution d'office et le versement du montant des travaux. Plutôt que la consignation d'une somme entre les mains du comptable public avant l'exécution d'office, l'amendement prévoit la réalisation des travaux, suivie du recouvrement de la dépense auprès des contrevenants. Cette dernière procédure est plus rapide et plus adaptée à des montants de travaux susceptibles d'être réglés par des particuliers. La consignation préalable relève davantage de dommages et de travaux importants. L'amendement proposé précise les conditions de mise en oeuvre de l'exécution d'office et, surtout, permet de mieux graduer la sanction administrative dans le temps, tout en préservant les droits du contrevenant à présenter des observations. Quel

la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés et le pouvoir de police associé.

autrement. Comme je le disais tout à l'heure au sénateur Chaize, il faut continuer à réfléchir à une mutualisation

fixe notamment les modalités de collectes sélectives et impose la séparation de certaines catégories de déchets, en particulier du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit réalisable sur le plan technique. Si la communauté de communes

Nos liens vont en souffrir

l'identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées. Il est également prévu que le maire puisse délivrer ces mêmes informations au responsable de la police municipale de sa commune. En contrepartie, le maire est tenu au secret. Quel est l'avis de la commission secret. Quel est l'avis de la commission ? radicalisation de certaines personnes- j'observe que le ministre de l'intérieur a diffusé, le 13 novembre 2018, une instruction enjoignant aux préfets de transmettre

Marie-Pierre de la Gontrie. Cet amendement vise essentiellement à aligner les pouvoirs de police des « agents de la Ville de Paris chargés d'un service de police », qui exercent actuellement les compétences de police municipale, sur le droit commun des agents de police municipale.

son histoire, les pouvoirs de police y sont essentiellement exercés par l'État, c'est-à-dire le préfet de police, et en partie seulement par le maire de Paris. Nous proposons aujourd'hui de faire entrer dans le droit commun

compte. Quel est l'avis de la commission ? À l'époque, certains, qui sont présents ici ce soir, avaient proposé un dispositif à peu près similaire, quoique

En effet, l'alignement des missions des agents de la Ville de Paris sur celles des agents de police municipale ne saurait se faire sans un alignement des conditions de recrutement et de formation. de formation. C'est pourquoi, par exception aux règles applicables à la fonction publique parisienne, nous estimons indispensable que le statut de ces agents soit défini par un décret en Conseil d'État. Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.

? Je le dis très clairement, le zèle des récents convertis vous pousse à déposer un amendement contre lequel vous auriez voté s'il avait été présenté voilà ne serait-ce que six mois.

explication de vote. Les Parisiens sont les citoyens français qui bénéficient le moins de la protection d'une police municipale.

attaquer. C'est tout de même la première fois, sous la VRépublique, qu'un Président de la République délaisse la région-capitale sur le plan des institutions. Le périmètre actuel de la préfecture de police ne correspond pas à la métropole du Grand Paris. Un certain nombre de réformes institutionnelles devaient être faites, mais on attend

à Paris. Avec Bertrand Delanoë, puis Anne Hidalgo, nous nous sommes nous aussi inscrits dans cette histoire, qui est l'histoire des rapports entre Paris et l'État.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Je vous invite, mes chers collègues, à vérifier que votre carte de vote est bien insérée dans votre terminal. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.

Je tenais à féliciter le rapporteur, qui est pour beaucoup

pas l'objectif. Il est de la responsabilité du maire, au titre de son pouvoir de police générale, de réglementer tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, en particulier en s'assurant de l'éclairage public. Il lui appartient donc, au cas par cas,

au premier rang desquelles le maire, de procéder à l'enlèvement des véhicules hors d'usage. Ainsi, le maire peut mettre en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation de remettre le véhicule en état et recourir à un expert automobile pour déterminer si le véhicule est réparable ou non.

système d'immatriculation des véhicules -utilisée par la police et la gendarmerie, et non un simple droit de transmission de ces informations, comme c'est le cas actuellement. La DGFiP pourrait ainsi procéder au recouvrement des avances sur frais et soulager, en termes de procédure et de financement, nos communes. Quel

Cet amendement nous paraît tout à fait satisfait par les dispositions du code de la route qui prévoient que les informations contenues dans le SIV sont communiquées, au moyen d'un accès direct, aux agents habilités de l'administration des finances publiques pour l'exercice de leurs compétences. Je vous demande donc de bien

est à M. Jérôme Durain. Sur proposition des rapporteurs, la commission des lois a adopté un nouvel article 15 dont le dispositif systématise l'information du maire par le parquet concernant les suites judiciaires et décisions de justice relatives aux infractions commises sur le territoire de la commune. Jusqu'à présent, cette information est transmise sur demande du maire.

celle des maires qui devront traiter les informations transmises. Enfin, il est nécessaire de préserver le respect des droits des personnes dont la condamnation ne nécessite pas systématiquement une information du maire de la commune. Pour ces proposons de supprimer les alinéas 1 et 2 de l'article 15 tout en en conservant l'alinéa 3. Il paraît en effet légitime que le maire soit informé des désordres qui se produisent sur le territoire de sa commune. L'extension de l'information des maires, à leur demande, aux suites judiciaires données aux infractions constatées par les agents de la police municipale paraît tout à fait justifiée.

par la police municipale. Une telle modification ne nous paraît cependant pas souhaitable, car elle risquerait d'entraîner un engorgement des parquets. Je note d'ailleurs que les maires, s'ils demandent à être informés des suites judiciaires données aux infractions ayant causé

est ainsi libellé : La parole est à M. Éric Gold. Cet amendement vise à prévoir l'interdiction du simple rappel à la loi, sauf accord de la victime, en cas d'infraction commise sur une personne dépositaire de l'autorité publique chargée d'une mission de service public ou sur une personne investie d'un mandat électif. Selon l'étude du Sénat sur la sécurité des maires récemment publiée, seulement 21 % des plaintes déposées par les maires ayant participé à l'étude ont abouti à une condamnation pénale des fautifs. On découvre ainsi que, dans 40 % des cas, les plaintes ne font l'objet d'aucune poursuite pénale. Dans cette dernière hypothèse, on pourrait avoir des mesures alternatives, comme des rappels à la loi ou des stages de citoyenneté. Les maires subissent aujourd'hui des atteintes physiques ou verbales que notre République ne saurait tolérer. Afin de restaurer leur autorité, il nous semble indispensable d'interdire le simple rappel à la loi en cas d'infraction commise sur leur personne dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions publique. Quel est l'avis de la commission ?

Il est souhaitable que la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par un élu victime d'un délit ne soit plus soumise, en l'absence de réponse du procureur de la République l'informant de son intention de ne pas engager les poursuites, à l'écoulement d'un délai de trois mois. Le délai de trois mois requis

en précisant que les conditions de recevabilité d'une constitution de partie civile, notamment le délai de trois mois, ne s'appliquent pas aux personnes dépositaires de l'autorité publique chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif public dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions. Quel est l'avis de la commission ?

Gold. L'étude du Sénat sur la sécurité des maires nous apprend que, dans les cas d'agression physique de maires, seulement 24 % des plaintes ont donné lieu à une condamnation pénale. On découvre aussi que, dans 16 % des cas, les plaintes font l'objet d'un classement sans suite. Cet amendement prévoit un dispositif correcteur. Dans le cas d'un délit contre un élu, le procureur serait désormais tenu de faire traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal, si et seulement si les conditions de la comparution immédiate sont remplies d'une part, que les charges réunies soient suffisantes, et, d'autre part, que l'affaire soit en état d'être jugée. Cet amendement prévoit une exception limitée au principe de l'opportunité des poursuites dans un cas très circonstancié, celui des délits contre une personne dépositaire de l'autorité publique chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif

prévoit de faire bénéficier de cette solution les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale y compris lorsque celui-ci ne fait pas partie du groupement de commandes, en lui permettant d'intervenir en leur nom et pour leur compte dans la passation, mais aussi l'exécution, de marchés publics destinés à répondre à leurs besoins. Dans cette perspective, l'EPCI intervient en tant que mandataire de ses communes membres, indépendamment des besoins qu'il pourrait avoir et des compétences qui lui ont été transférées, mais sous réserve que ses statuts le prévoient. Si ce dispositif est intéressant en ce qu'il permet d'optimiser la dépense en mutualisant une fonction support entre communes membres d'un EPCI, il n'en demeure pas moins que cette nouvelle mission peut constituer une charge pour l'intercommunalité, qui doit pouvoir décider, avec ses communes membres, si elle souhaite l'assumer à titre gracieux ou pas. Actuellement, le groupement de commandes n'est possible qu'en matière de passation de marchés. De surcroît, il donne lieu à une convention qui définit les modalités de fonctionnement du groupement. La modification proposée n'ôte pas la possibilité de conclure une convention à titre gracieux, mais laisse le choix à l'EPCI et à ses communes membres d'en décider.

de donner aux EPCI, seuls ou regroupés, la latitude d'élaborer, avec l'ensemble des acteurs du territoire, une charte de développement commercial,

Le rapport au Parlement de février 2012 sur les conséquences de la création d'une agence de financement des collectivités locales a conduit à la création du groupe Agence France locale par la loi du 26 juillet 2013. Construit sur le modèle des agences de financement des collectivités locales nordiques, le groupe Agence France locale est reconnu comme fédérateur pour les collectivités locales. Plus de 310 collectivités locales, régions, départements, métropoles, communautés et communes de toutes tailles, sont aujourd'hui actionnaires de la société mère du groupe, la société territoriale. Ce modèle est suivi par des investisseurs financiers du monde entier. L'agence a déjà accordé plus de 2,8 milliards d'euros de crédits à ses membres. Elle a commencé ses activités de prêt en avril 2015. Ses membres peuvent ainsi financer des investissements, à travers leurs budgets principaux ou leurs budgets annexes. Cependant, concernant les EPCI, seuls ceux à fiscalité propre peuvent aujourd'hui devenir actionnaires de l'Agence France locale. Or, dans de nombreux cas, la compétence s'exerce par le biais d'un syndicat. Ainsi, en l'état actuel des textes, une même compétence peut, lorsqu'elle est exercée un budget annexe, bénéficier des financements de l'AFL, alors que ce n'est pas possible lorsqu'elle est exercée par un syndicat. C'est pourquoi il convient de corriger cette anomalie et de permettre auxdits syndicats de pouvoir bénéficier des services du groupe, en élargissant la base potentielle des actionnaires de protection, cet élargissement, une fois autorisé par la loi, sera encadré dans les statuts des deux sociétés du groupe et strictement décrit dans sa documentation, afin de préserver la rigueur de la sélection des nouveaux actionnaires,

d'une part, il vise à élargir les catégories de personnes morales habilitées à devenir actionnaires de l'Agence France locale aux groupements de collectivités locales et aux établissements publics locaux, corrigeant par là même une anomalie législative de premier ordre qui les avait jusqu'ici injustement exclus du dispositif d'autre part, il tend à encadrer par voie réglementaire l'extension de la base potentielle des actionnaires, afin que soient précisées les modalités d'application concrète, notamment les conditions d'adhésion et les seuils applicables à leur situation financière et à leur niveau d'endettement.

À titre d'illustration, en 2018, l'agence a couvert 5,1 % des crédits à long terme des collectivités, contre 2,7 % en 2017.

monsieur le ministre,

Pour les conseillers municipaux qui ne sont pas délégués communautaires, le fonctionnement et les décisions de l'intercommunalité apparaissent souvent bien lointains. Certes, plusieurs mécanismes d'information sont d'ores et déjà prévus par la loi, nous en avons déjà renforcé quelques-uns au début de la discussion de ce texte. Il me semble toutefois primordial de remettre de l'humain et du débat là où la transmission de rapports et de notes techniques ne suffit pas toujours à éclairer

d'une part, lever les difficultés que rencontrent les EPCI pour justifier de leurs besoins afin de participer aux groupements de commandes ; d'autre part, inciter à la mutualisation des achats et aux économies d'échelle permises par ces groupements.

Nous avons engagé ce débat avec l'idée, développée tant par le Gouvernement que par les rapporteurs, de supprimer les irritants et d'aller, pour reprendre la formule d'un des rapporteurs, vers une « intercommunalité heureuse

que les communes pourront transférer à la carte ce qu'elles souhaitent à l'intercommunalité, l'article 17 prévoit que les intercommunalités seront libres de subdéléguer au département et à la région.

à rendre l'action publique plus efficiente, en prenant en compte la diversité des territoires et le fait que la loi NOTRe et un certain nombre d'autres lois, mais aussi, parfois, la gouvernance des établissements

la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions à toute autre collectivité territoriale. Le dispositif

qu'elle soit. Lorsque la commune peut exercer la compétence, il n'y a pas de raison que la communauté de communes l'exerce. Nous prévoyons donc la possibilité de restituer des compétences. Il faudra d'ailleurs que nous traitions la question de la neutralité financière, pour la communauté de communes, de ces restitutions de compétences à la commune.

et si par ailleurs le département ou la région le désirent, qu'une convention entre le département et la région permette à cette compétence d'être exercée au meilleur niveau, qui n'est alors pas celui de la communauté de communes. Jusqu'à présent, c'est interdit pour une raison de principe très simple : on considère que la communauté de communes n'a pas la compétence de sa compétence et qu'elle ne peut déléguer à autrui ses compétences,

Il n'y a rien à craindre de ce mouvement, pour la simple et bonne raison qu'il faut, d'un côté, que la communauté de communes soit d'accord, et, de l'autre, que le département ou la région soient également d'accord. Je ne connais pas de communauté de communes, monsieur le ministre, qui aurait l'intention de se dépouiller de l'intégralité de ses compétences. C'est une absurdité que d'imaginer cela

les statuts de la communauté de communes. Or, vous le savez bien, ces statuts sont adoptés à une majorité qualifiée : soit les deux tiers des voix, représentant au moins 50 % de la population

la volonté des communes. Toute l'habileté du président Philippe Bas ne m'empêchera pas de lui dire qu'il plaide en fait pour la confusion des pouvoirs

Prenons un seul exemple : la compétence économique. Que de débats ici pour dire qu'elle relève des régions, en lien avec l'intercommunalité ! Je connais des départements qui ne l'ont toujours pas digéré et qui veulent

La perspective de la décentralisation était de répartir les compétences entre trois blocs : à la commune, la proximité et l'urbanisme ; au département, la solidarité ; à la région, l'économie. Entre-temps est arrivé l'échelon intercommunal. ici, vous proposez de faire de la différenciation sans maîtriser aucunement les conséquences de cette dernière. En effet, la différenciation se fera à la carte, différemment en fonction des périmètres territoriaux,

des transferts de compétences ou qu'il faut les évaluer. Je dis simplement que le système mis en place par la commission est beaucoup trop simple et trop simpliste. C'est la difficulté : il n'est pas assez encadré

On a parlé tout à l'heure de la création d'une police municipale à Paris- mesure qui faisait partie du texte sur le statut de Paris -et des aménagements métropolitains. Vous avez vous-mêmes préconisé la création de cette métropole. Vous affirmez aujourd'hui, avec une grande solennité,

cher Jean-Pierre Sueur, qui exerce en plein ses compétences, puisque tout cela relève d'un montage artificiel- je le dis très clairement, car c'est pour ça que nous y sommes opposés -, d'une répartition entre

il est paradoxal de nous renvoyer à la question de l'accord de la commune s'agissant de l'eau et l'assainissement quand, à la surprise générale, alors même que vous aviez voté à l'unanimité le texte, vous avez refusé de rendre facultative

la notion de proximité. Pour avoir fait le tour d'à peu près tous les départements et pour avoir vu comment s'étaient constitués les schémas départementaux de coopération intercommunale,

objectif de servir l'efficacité de l'action publique, et non de tricoter, de détricoter ou de conserver comme un vase sacré je ne sais quelle structure et quelle compétence

Cartron. Cet article permet aux EPCI à fiscalité propre de déléguer leurs compétences à un département ou à une région. M. le ministre l'a souligné, ce système de délégation ascendante, sous couvert d'un assouplissement juridique, ne va pas dans le sens de la ligne directrice de ce projet de loi : au lieu d'apporter les correctifs nécessaires,

En effet, si à ce jour, conformément à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, une commune ou toute autre collectivité territoriale peut déléguer sa compétence à un EPCI à fiscalité propre, l'inverse n'est pas prévu par la loi. Il n'est pas non plus envisageable pour un EPCI à fiscalité propre de déléguer l'exercice d'une de ses compétences à une structure syndicale. La délégation de compétence permet pourtant de confier l'exercice d'une compétence d'attribution à une collectivité ou à un EPCI qui dispose de l'expérience, de l'expérience, des moyens, mais également de la volonté de l'exercer par la simple voie contractuelle. Ce mode d'exercice de la compétence est davantage pérenne et plus sécurisé que les simples conventions de gestion ou de prestations de services. L'élargissement du champ d'application de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales pourrait, d'une part, être synonyme de lisibilité